Monsieur le président,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

il est d'usage, en nouvelle lecture, de ne pas refaire une présentation des grandes mesures d'un texte déjà débattu en première lecture. Aujourd'hui, l'exercice revêt un caractère particulier. Comme l'ai déjà dit ici je regrette que les circonstances de la première lecture ne nous aient pas permis d'aller au bout de l'examen de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS). J'aurais naturellement préféré que la situation soit différente, mais nous n'étions pas prêts, à ce moment-là. J'espère, à présent, que nous aurons le débat que ce texte mérite. De nouvelles annonces ont été présentées, la semaine dernière, pour investir dans l'hôpital et soutenir la transformation engagée par Ma santé 2022- une transformation que je sais soutenue par beaucoup d'entre vous. Il s'agit de redonner de la souplesse et des marges de manoeuvre pour améliorer le quotidien des hospitaliers et accélérer la transformation. Nous avons eu, vous avez eu, l'occasion de dire les difficultés que traverse l'hôpital, notamment public. La mobilisation du 14 novembre dernier a montré l'épuisement, voire la colère, des personnels soignants comme non soignants. Ces mesures s'articulent autour de trois axes principaux. Le premier vise à restaurer l'attractivité des métiers et à fidéliser les soignants. Il s'agit donc de mieux reconnaître les personnels en accompagnant les débuts de carrière pour restaurer la capacité des hôpitaux ensuite concentrer l'effort sur la revalorisation des métiers en tensions, qu'il s'agisse de tensions territoriales, comme à Paris et dans la petite couronne, où une prime de 800 euros sera attribuée aux hospitaliers, ou bien de tensions sectorielles, notamment pour le métier d'aide-soignant. exerçant dans les services qui prennent en charge les personnes âgées bénéficieront ainsi de la prime assistant de soins en gérontologie. Par ailleurs, les aides-soignants pourront désormais accéder, dans le cadre d'un grade de fin de carrière, à la catégorie B. Il nous faut également récompenser l'investissement et l'engagement collectifs avec la création d'une prime d'intéressement, à la main des responsables, de manière à pouvoir récompenser des équipes qui s'engagent sur le terrain autour de projets relatifs à la qualité du service ou à la transformation.

L'hôpital public a connu des évolutions majeures dans son organisation, qui ont parfois donné aux équipes le sentiment d'une mise à l'écart de la prise de décision et d'une perte de sens. La stratégie de transformation Ma santé 2022 vise à renforcer le dialogue et le sens du collectif au sein des hôpitaux. Pour ce faire, le personnel soignant sera mieux intégré à la gouvernance des hôpitaux et le management de proximité sera renforcé et valorisé. Des mesures de simplification du fonctionnement quotidien seront aussi prévues, notamment en termes de formalités de recrutement ou bien de protocole de coopération décentralisée entre les professionnels au sein d'un établissement. Enfin, des mesures seront prises pour lutter contre l'intérim médical, dont vous savez qu'il s'est déployé depuis plusieurs années dans des conditions devenues insupportables pour les équipes ayant la charge d'assurer la continuité du fonctionnement des hôpitaux. Notre troisième axe consiste à réinvestir l'hôpital public en lui donnant des moyens nouveaux et de la visibilité dans le temps. Les tarifs hospitaliers seront en hausse- seront en hausse- -de 0,2 % jusqu'à la fin du quinquennat après la première campagne positive exceptionnelle de 2019, interrompant ainsi dix années de baisses successives. L'investissement du quotidien sera une priorité. Il s'agit de permettre aux hôpitaux d'acheter du matériel indispensable pour le travail des soignants dans leur quotidien. En 2020, 150 millions d'euros seront donc fléchés vers l'investissement courant, au lieu d'être engagés dans de nouveaux grands projets immobiliers, pour répondre au besoin actuel le plus fort. Cet effort de 150 millions d'euros sera reconduit en 2021 et en 2022. À partir de 2020, 10 milliards d'euros de dettes seront repris aux hôpitaux en trois ans afin d'alléger les charges des établissements. Cette décision de rupture permettra aux hôpitaux de réduire leur déficit et de retrouver rapidement les moyens d'investir et de se moderniser. Ce PLFSS porte, au-delà de l'Ondam, un ensemble de mesures dont chacun peut être fier. Je pense en particulier au congé de proche aidant, à la lutte contre les ruptures d'approvisionnement de médicaments, à la création du fonds d'indemnisation des victimes des produits phytosanitaires,

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission des affaires sociales, monsieur le rapporteur général, mesdames, messieurs les rapporteurs de branches, mesdames, messieurs les sénateurs,

Nous savons l'opposition renouvelée du Sénat et je préfère dire d'emblée- peut-être pour gagner du temps lors des explications de vote -que le Gouvernement restera sur sa position en émettant un avis défavorable sur les amendements adoptés par la commission des affaires sociales tendant à la suppression de cet article.

Les échanges que nous avons eus cet automne soulignent la nécessité d'avoir prochainement un débat sur l'avenir des relations entre l'État et la sécurité sociale. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Je souhaite également insister sur l'article 7 et l'obligation pour une entreprise d'avoir conclu un accord d'intéressement pour pouvoir bénéficier de l'exonération de la prime exceptionnelle. Cette mesure, qui s'inscrit en cohérence avec la politique du Gouvernement- notamment depuis la loi Pacte -de promouvoir l'intéressement et la participation dans les entreprises, permet de renforcer le pouvoir des salariés de manière pérenne durant toute la durée de l'accord d'intéressement et pas uniquement pour la seule année du versement de la prime exceptionnelle.

J'en viens maintenant aux équilibres financiers de ce texte que les mesures sur l'hôpital ne remettent pas fondamentalement en cause, puisque nous assumons des dépenses nouvelles de 3 milliards d'euros sur trois ans. Celles-ci doivent permettre d'offrir aux soignants des conditions de travail satisfaisantes en dégageant des moyens supplémentaires dans la durée. Elles permettront également aux établissements d'investir et de se transformer. Ces dépenses supplémentaires seront intégrées à la trajectoire des finances publiques présentée dans la loi de programmation des finances publiques au premier semestre 2020. Ce texte précisera les orientations du Gouvernement en matière de recettes et de dépenses publiques pour les prochaines années. Un mot, pour terminer, sur la reprise de dette des hôpitaux dont vous aurez à connaître dans un projet de loi qui sera déposé début 2020. L'allégement de la dette de 10 milliards d'euros en trois ans est d'abord un fait historique et une mesure exceptionnelle : cela va permettre de dégager des marges de manoeuvre pour les hôpitaux afin qu'ils puissent réduire leur déficit et investir. Au bout de trois ans, la reprise de dette va alléger la charge des hôpitaux de 800 millions à 1 milliard d'euros par an, en fonction de la dette reprise et des taux d'intérêt afférents. Il s'agit d'une bouffée d'oxygène bienvenue. bienvenue. Cette reprise de dette ne se traduira pas par une augmentation parallèle de la dette publique, dans la mesure où la dette des hôpitaux y est déjà comptabilisée, au regard des instances et de nos partenaires européens. Nous serons vigilants, aux côtés des établissements, pour que les marges de manoeuvre supplémentaires dégagées contribuent non pas à recréer de la dette, mais bien à accélérer la transformation de l'hôpital public que le plan Ma santé 2022 avait engagée et qui doit être mise en oeuvre jusqu'à son terme. Nous assumons ces choix budgétaires. Notre rythme d'ajustement budgétaire est certes différent de celui qui était envisagé en 2017, mais il tient compte à la fois du ralentissement économique mondial, des difficultés sociales que traverse notre pays et des priorités que nous assumons de financer. de financer. Ce texte s'inscrit dans la continuité de la politique que nous menons depuis plus de deux ans, à la fois pour baisser les impôts et pour soutenir le pouvoir d'achat des Français. Il est en cohérence avec nos objectifs. Il nous permet d'aller plus loin et d'apporter des réponses à la

que nous ne disposions d'aucun élément chiffré. De même, la commission mixte paritaire, convoquée la veille de l'annonce du plan gouvernemental, a rapidement constaté son désaccord politique et le caractère un peu vain de l'exercice dans ce contexte particulier.

a repris l'amendement de la commission tendant à préciser explicitement l'obligation faite au distributeur de mentionner au patient concerné que le dispositif médical remis en bon état d'usage est bien le même que celui qui elle a repris l'amendement de la commission visant à étendre à tous les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur l'obligation d'information des autorités de la suspension ou de l'arrêt de commercialisation par les établissements pharmaceutiques.

à l'obligation de déclaration relative aux disponibilités d'accueil de l'assistant maternel ne puisse constituer un motif de suspension de l'agrément ou le seul motif de son retrait. Mme Doineau En outre, l'Assemblée nationale a intégré, à l'article 59 et dans divers articles récapitulatifs, la hausse de l'Ondam de 300 millions d'euros correspondant à la première année du plan Hôpital annoncé par le Gouvernement. Aucune mesure de hausse de recettes ou de baisse de dépenses n'ayant accompagné ce plan, ces 300 millions d'euros augmentent le déficit de la sécurité sociale pour 2020.

Surtout, il est inquiétant de constater que le rapport annexé au PLFSS prévoit désormais des comptes en déficit au moins jusqu'en 2023

malgré une prévision de recettes assez optimiste aux yeux de la commission. Une telle situation ne fait que renforcer plusieurs des analyses exprimées par le Sénat. Je pense en particulier à la nécessité de renoncer au principe de non-compensation. En effet, on ne saurait demander à la sécurité sociale de financer toujours plus de dépenses de nature assurantielle tout en la privant de ressources au nom de politiques gouvernementales d'augmentation du pouvoir d'achat. Cela n'aboutira qu'à créer toujours plus de déficits et à repousser toujours plus loin les perspectives d'en finir avec la dette sociale. Il me semble, mes chers collègues, que c'est le rôle du Sénat que de l'affirmer haut et fort, clairement, et de l'inscrire dans un texte que nous voterons. Permettez-moi un texte que nous voterons. Permettez-moi de citer un courrier que les deux rapporteurs généraux des commissions des affaires sociales de l'Assemblée nationale et du Sénat ont récemment reçu du Premier ministre, en réponse à leur interpellation sur le sujet des non-compensations. M. Édouard Philippe nous donne l'assurance « qu'aucun autre transfert ou non-compensation n'est envisagé par le Gouvernement pour 2021 ou 2022 ». Nous en

et de la doctrine des relations financières entre l'État et la sécurité sociale, ce que permettra le prochain projet de loi de programmation des finances publiques ». Madame la ministre, monsieur le secrétaire d'État, nous aurons donc l'occasion de poursuivre ce débat dès le printemps prochain. Cette nouvelle lecture devrait nous permettre d'aborder des articles que nous n'avons pas examinés en séance publique en première lecture. La commission affirmera ainsi sa volonté de réindexer, dès 2020, l'ensemble des prestations et allocations de sécurité sociale sur l'inflation, qu'il s'agisse notamment des allocations familiales, de l'allocation aux adultes handicapés ou des pensions de retraite. À cet égard, la contrainte de « l'entonnoir » ne permettra au Sénat que de livrer une vision tronquée de ses propositions, puisque d'importantes mesures d'économies, comme le recul de l'âge légal de départ à la retraite, ne pourront être présentées dans le cadre de cette nouvelle lecture.

En tant que rapporteur général, je serai, bien entendu, le fidèle interprète des votes de la commission, laquelle a estimé insuffisante la hausse de 300 millions d'euros par rapport à la première lecture. en introduction de nos débats, il me semble important de rappeler ce qu'est l'Ondam. Ce n'est pas un taux- de 2,3 % ou 2,45 %-, c'est un montant de dépenses publiques,

rapport à 2019. Je pense qu'aucun autre budget public n'affiche une telle augmentation, très nettement supérieure à la croissance de la richesse nationale, année après année.

et une chose légitime, de dire que, ponctuellement, le geste en faveur des hôpitaux aurait pu être un peu plus fort. C'en serait une autre de nier la nécessité même de contrôler la hausse tendancielle des dépenses de santé de plus de 4 % par an et que nous serions très vite incapables de financer.

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, lors de l'examen en première lecture du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, notre groupe avait déjà déposé une motion tendant à l'irrecevabilité constitutionnelle, au motif que les exonérations massives de cotisations sociales et leur non-compensation intégrale par l'État remettent en question l'autonomie financière de la sécurité sociale. Nous récidivons pour cette nouvelle lecture, car, si le non-respect de la loi Veil du 25 juillet 1994 est toujours de mise, vous remettez maintenant en cause l'organisation des travaux parlementaires telle que prévue à l'article 47-1 de la Constitution. Deux motifs graves qui justifient cette motion d'irrecevabilité constitutionnelle. Madame la ministre, monsieur le secrétaire d'État, je le dis avec solennité : que cherche le Gouvernement en refusant de voir la réalité de terrain ? Les mesures que vous avez annoncées avec le Premier ministre ne font pas le compte. Et même si ce plan Investir dans l'hôpital public est une première victoire des personnels en lutte, leur colère ne retombe pas. Fort justement, car les mesures demeurent largement insuffisantes par rapport aux besoins en matière de santé. D'ailleurs, aujourd'hui même est une journée d'initiatives locales dans les établissements et autour, avant la mobilisation du 17 décembre et, auparavant, celle du 5 décembre, qui promet d'être de grande ampleur avec une participation forte du monde de la santé.

Nous avons assisté en direct, ici, au Sénat, en première lecture du PLFSS, à vos atermoiements et au peu de cas que vous faites de notre Haute Assemblée. Ce n'est pas un procès d'intention, c'est une réalité que chacune et chacun peut vérifier en suivant la retransmission de nos travaux. La publication, l'avant-veille de l'examen du budget de la sécurité sociale, d'un article dans le faisant état de la préparation d'un « plan ambitieux pour l'hôpital » a profondément entaché l'examen en première lecture du budget de la sécurité sociale. vous nous avez affirmé, aux côtés du secrétaire d'État Dussopt, que ces fuites dans la presse ne venaient pas de vous et que vous respectiez trop les parlementaires que nous sommes pour ne pas nous informer de modifications qui pourraient remettre en cause le budget que nous examinions. Mais cela, c'était deux jours avant la formidable mobilisation des professionnels de santé toutes catégories confondues, après une grève de plus de huit mois. Alors que le Sénat poursuivait la discussion du budget de la sécurité sociale, le Président de la République annonçait bien un « plan conséquent pour l'hôpital public ». Tant pis pour la représentation nationale qui discutait d'un texte obsolète et, de fait, d'un budget insincère. Nous avons alors décidé, à l'unanimité, d'interrompre nos débats et de repousser l'examen du PLFSS 2020 à la nouvelle lecture, car il s'agissait d'une véritable mascarade démocratique. Comment croire que vous n'avez rien anticipé ? Comment croire les propos que vous avez tenus devant la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, affirmant que vous n'étiez pas prêts en première lecture ? Pas prêts, après plus de huit mois de mobilisation des hôpitaux ? Soyons sérieux ! La réalité, c'est que vous avez attendu de voir le niveau de la mobilisation des personnels hospitaliers du 14 novembre pour décider de la taille de l'enveloppe de votre plan pour l'hôpital. Ce plan Investir dans l'hôpital public est donc le quatrième plan d'urgence en quatorze mois pour l'hôpital. Il vient après le plan Ma santé 2022, présenté en septembre 2018, et voté par le le Parlement ; après les mesures pour les urgences annoncées en juillet 2019 ; et après le plan d'urgence de septembre dernier. Finalement, je me demande si s'adresser à vous, madame la ministre, revient à s'adresser à la ministre de la santé ou à la ministre de la planification

faut-il rappeler ici, mes chers collègues, que le Gouvernement avait initialement prévu de priver les hôpitaux publics de 1 milliard d'euros en 2020 ? Donc, si je calcule bien, avec vos largesses, vous le privez tout de même de 700 millions d'euros

soit 5 milliards d'euros de plus. Malgré le niveau de colère et de mobilisation justifié des personnels, vous refusez de débloquer les moyens indispensables pour répondre aux besoins de santé. Il s'agit bien d'un marché de dupes, car le relèvement de l'Ondam pour 2020, obtenu de haute lutte, est au-dessous du niveau de l'Ondam de l'an dernier, qui était de 2,5 %. Vous annoncez des moyens supplémentaires, mais vous maintenez la compression des dépenses de santé de l'hôpital public. Dans une tribune publiée mercredi 13 novembre dans la presse, près de 2 000 professionnels de santé en pédiatrie se sont élevés contre le manque de moyens dans les hôpitaux, notamment dans les services où sont soignés les enfants. Que répondez-vous au professeur Rémi Salomon, chef de service pédiatrie de l'hôpital Necker, quand il dénonce : « alors alors que l'épidémie de bronchiolite débute, on est obligés de transférer des enfants en dehors des hôpitaux parisiens » ? Tout le monde a bien conscience qu'il s'agit d'une prise de risque pour ces petits patients. À l'écoute de ce témoignage et à la lecture de cette tribune, votre plan d'urgence devrait comporter des ouvertures immédiates de lits, surtout quand on sait que 100 000 d'entre eux ont été fermés en vingt ans. Eh bien, pas du tout : vous persistez et vous signez dans vos choix mortifères pour l'hôpital. La réalité, c'est que vous ne répondez à aucune des revendications fondamentales des personnels qui sont attachés à l'hôpital et qui veulent des moyens réels pour améliorer la qualité des soins de leurs patients. À l'exigence d'une augmentation de 300 euros par mois des salaires, vous répondez par une prime catégorielle pour l'Île-de-France de 800 euros pour 40 000 infirmières et aides-soignantes. Prime qui ne prend pas en compte le vécu de ces professionnels sur l'ensemble du territoire et pas seulement en Île-de-France- 800 euros, c'est 66 euros par mois, soit moins que le coût d'un pass Navigo De plus, une prime n'entre pas dans le calcul de la retraite, contrairement au salaire. Voilà une manoeuvre grossière pour essayer d'affaiblir la mobilisation en cherchant à opposer les personnels entre eux,

Vous poursuivez sans ciller les fermetures de services, et d'hôpitaux, sous le vocable de « regroupement », malgré l'aggravation des déserts médicaux. La France dépenserait trop pour la santé, contrairement à ses voisins, dites-vous ! Des économistes de la santé contredisent cette affirmation.

Votre leitmotiv est qu'il n'y a pas d'argent magique et que, par conséquent, vous devez respecter les contraintes budgétaires. Mais, madame la ministre, faites cesser les exonérations de cotisations sociales et vous aurez de nouvelles recettes, récoltée s'élevant à 66,4 milliards d'euros pour 2020. Si vous cherchez des cotisants, sachez que nous avons la chance d'avoir, en France, la première fortune du monde, évaluée à 109,5 milliards d'euros, en la personne de M. Bernard Arnault, patron de LVMH ! Madame la ministre, comment Madame la ministre, comment ne pas dénoncer le fait que ces allégements et exonérations dépassent le montant des recettes de la branche famille ?

J'ai dit au début de mon propos que votre plan « Investir pour l'hôpital public » était un marché de dupes, mais c'est, de surcroît, le bal des hypocrites ! Si vous renonciez ne serait-ce qu'à un tiers de ces exonérations, vous dégageriez 20 milliards d'euros pour l'hôpital, de quoi répondre à la crise aiguë qu'il connaît aujourd'hui.

la reprise sera conditionnée à l'adoption de plans de suppressions de postes ? Quel hôpital aura vos faveurs, alors que six hôpitaux sur dix sont en déficit et qu'un tiers des établissements publics, soit 319 hôpitaux, 19 centres hospitaliers régionaux (CHR) et en situation de surendettement ? On ne peut tergiverser : il est urgent d'assurer le financement d'investissements en faveur des établissements médico-sociaux et de santé, donc de revenir aux prêts à taux zéro. taux zéro. Mes chers collègues, le contenu du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 dont nous discutons en nouvelle lecture et les conditions d'examen dans lesquelles nous nous retrouvons ce matin, avec une injonction implicite de légiférer très vite, contreviennent aux principes constitutionnels.

Par ailleurs, il importe que le Sénat puisse se prononcer sur ce PLFSS et donner ainsi sa propre vision- c'est ce que je disais sur les finances sociales. En conséquence, la commission émet un avis défavorable

des objectifs qu'ils ont défendus pour une nouvelle politique de santé. Nous avions d'ailleurs voté une motion analogue en première lecture. Mais nous pensons, aujourd'hui, qu'il faut débattre, cela pour au moins deux raisons. Le plan Hôpital est maintenant connu ; le nouvel Ondam et la majoration de 200 millions plus 100 millions d'euros sont parfaitement identifiés. Et nous devons avoir l'occasion de dire soit tout le bien,

d'image dans l'opinion publique, à interrompre cette discussion. Nous ne voterons donc pas la motion qui vient d'être présentée.

projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020. Ainsi le groupe RDSE ne votera-t-il pas non plus cette motion.

Je rappelle également que l'avis de la commission est défavorable et que l'avis du Gouvernement est défavorable. En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.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

Le 14 novembre dernier, les organisations syndicales et les collectifs des personnels de la santé étaient en grève. Devant l'ampleur de la mobilisation des blouses blanches, le Président de la République a senti la nécessité d'annoncer un « plan fort » pour l'hôpital.

Nous espérions qu'enfin vous aviez compris qu'il fallait stopper la réduction des dépenses publiques. Mais nous avons vite déchanté. En définitive, il s'agissait davantage de tenter d'endiguer le mouvement social, en lâchant un peu de lest,

alors que les organisations syndicales estiment les besoins à 5 milliards d'euros par an ! Même la Fédération hospitalière de France réclame 1 milliard d'euros par an pour réinvestir.

Vous annoncez une prime de 800 euros annuels, soit 66 euros par mois, pour les infirmières et infirmiers, ainsi que pour les aides-soignantes et les aides-soignants gagnant moins de 1 900 euros. Madame la ministre, prime ne vaut pas salaire ! Les collectifs Inter-Urgences exigent 300 euros de revalorisation salariale par mois pour tous les personnels médicaux et paramédicaux. Vous avez préféré cibler les personnels d'Île-de-France alors que l'ensemble du territoire est concerné, tentant ainsi de diviser les personnels entre eux. à la reprise de 10 milliards d'euros de la dette des hôpitaux, elle est suspendue à une nouvelle loi qui en fixera les conditions. Mais l'essentiel est déjà connu : les établissements devront solliciter une demande de reprise partielle de dettes, qui se fera en échange d'un engagement contractuel avec l'État. Vous appliquez la stratégie que le FMI applique aux pays en crise : annulation partielle de dettes en échange d'une politique d'austérité, en lieu et place d'un vaste plan d'investissements pourtant indispensable.

Je pourrais vous parler de ma région, des centaines de personnels en grève ou mobilisés au centre hospitalier de Douai comme à ceux de Tourcoing, de Valenciennes, de Lille, de Seclin. Je pourrais vous parler de celui de Lens, où les urgences sont en grève depuis des semaines, de bien d'autres encore. entendre la même colère et les mêmes revendications, auxquelles votre plan ne répond pas : des moyens supplémentaires pour ouvrir des lits, embaucher du personnel et revaloriser les salaires. Vous préférez continuer à faire des cadeaux aux plus riches et faire peser l'austérité sur les plus fragiles. Qu'il s'agisse de la désindexation des pensions de retraite et des prestations familiales, de la suppression de la majoration des indemnités journalières pour les parents de familles nombreuses ou de ou de l'absence de mesures pour les services d'aide et d'accompagnement à domicile, votre obstination ne fait que réduire le pouvoir d'achat du plus grand nombre. Madame la ministre, nous vous appelons à tenir compte des propositions alternatives que nous avons construites avec nos collègues députés du groupe de

Si vous aviez pris le temps de le lire, vous auriez vu qu'y figurent des propositions qui sont, aujourd'hui, les principales revendications des personnels mobilisés : l'augmentation du budget de la santé à hauteur de l'évolution naturelle des dépenses, la suppression de la taxe sur les salaires, l'instauration d'un moratoire contre les fermetures de lits, de services et d'établissements ou la redéfinition des missions des hôpitaux de proximité. Madame la ministre, écoutez les personnels qui se mobilisent, et écoutez la représentation parlementaire, quand bien même elle est dans l'opposition ! Cela vous éviterait de défendre un PLFSS caduc, car en dehors de la vraie vie ! La parole

nous sommes réunis pour examiner en nouvelle lecture le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, après avoir rejeté le texte en première lecture, dans l'attente des annonces du Gouvernement en faveur de l'hôpital public. Ce plan d'urgence, annoncé le 20 novembre dernier, est l'expression d'un effort particulier pour aider le secteur hospitalier à se remettre à flot. Il s'agit non pas, comme certains le diront, de mesures anecdotiques ou d'un simple saupoudrage, mais d'un engagement fort du Gouvernement, qui démontre sa capacité d'écoute et sa réactivité. Parmi ces engagements, la reprise d'un tiers de la dette du secteur représente un allégement de 10 milliards d'euros sur trois ans pour le budget des hôpitaux. de faciliter les carrières du personnel soignant et de renforcer l'attractivité de ces métiers essentiels que sont ceux d'infirmier et d'aide-soignant, le Gouvernement prévoit une revalorisation des rémunérations et du cadre de travail. La prime d'exercice territorial sera augmentée et étendue, et le personnel hospitalier travaillant en région parisienne bénéficiera d'une nouvelle prime annuelle. Dans l'idéal, cette prime devrait pouvoir profiter à l'ensemble des soignants, en tout point du territoire, mais nous sommes conscients des contraintes budgétaires qui obligent à de tels arbitrages. D'autres mesures suivront pour réformer le statut du médecin à l'hôpital et moderniser la gouvernance hospitalière. Nous soutiendrons l'amendement du Gouvernement visant à encadrer le travail intérimaire et à renforcer le contrôle des rémunérations et des temps de travail. L'objectif national de dépenses d'assurance maladie, inscrit à l'article 59 du présent texte, est relevé à hauteur de 2,45 % pour 2020. Cela représente une rallonge budgétaire de 300 millions d'euros dès l'année prochaine pour les établissements de santé. Suivront d'autres moyens, échelonnés sur trois ans, pour un total de 1,5 milliard d'euros. En complément, 150 millions d'euros seront directement alloués aux équipes soignantes pour financer les dépenses courantes, comme l'achat de nouveaux matériels. Nous l'avions dit en première lecture : notre groupe soutient le texte du Gouvernement et les nombreuses avancées qu'il contient. Madame la ministre, nous comprenons votre choix de faire porter à la sécurité sociale le poids des mesures sociales mises en oeuvre par l'État. Il fallait, par des réponses d'urgence et de moyen terme, apaiser les tensions qui traversaient notre pays sans pour autant pénaliser la France au regard de ses engagements européens. Notre seul désaveu porte sur votre choix de reconduire en 2020 la sous-revalorisation des prestations sociales à hauteur de 0,3 % de l'inflation. Les plus faibles retraites sont épargnées, mais le pouvoir d'achat des ménages les plus fragiles et des classes moyennes est pénalisé- nous le regrettons.

L'indemnisation du congé de proche aidant, à l'article 45, permettra aux salariés, sans condition d'ancienneté, de consacrer trois mois à un proche sur l'ensemble de leur carrière. Il s'agit d'une deuxième étape importante, après celle de la création de ce congé en application de la loi du 28 décembre 2015 ; 8 millions de personnes, en France, pourraient en bénéficier. Nous ne pouvons que saluer la création d'un fonds d'indemnisation pour les victimes de maladies professionnelles liées à l'utilisation de produits phytosanitaires, prévue à l'article 46. Nous sommes favorables à une couverture la plus complète possible des victimes.

Il est important de maintenir de telles obligations de stock sur l'ensemble de ces médicaments, et non uniquement sur ceux pour lesquels il n'existe pas d'alternative thérapeutique, afin de permettre au médecin de prescrire librement le remède le plus adapté à son patient. Parmi les mesures importantes du texte, je citerai également : la réforme du financement de la psychiatrie et des hôpitaux de proximité ; la prise en charge des cotisations sociales des jeunes médecins s'installant en zone sous-dense la création d'un droit au transport et à l'hébergement pour les femmes enceintes les plus éloignées des maternités. Ces mesures contribueront à réduire les inégalités territoriales d'accès à la santé et aux soins.

sur nos débats lors de la première lecture de ce PLFSS, que je pourrais qualifier de « grand-guignolesque » si les conditions de son examen n'étaient pas si graves pour nos institutions. Très juste ! Madame la ministre, monsieur le secrétaire d'État, je tiens à vous le dire solennellement

un tel mépris pour la représentation nationale. Le Gouvernement a en effet cherché à donner un rôle totalement factice au Sénat, le laissant délibérer sur un texte frappé d'emblée de caducité et d'insincérité. Je réitère la mise en garde que j'avais faite lors de mon intervention en première lecture : à trop vouloir se passer du Parlement et des corps intermédiaires, le Gouvernement finira par se face aux mouvements sociaux en cours ou à venir. Un tel face-à-face est dangereux, soumis au risque inhérent aux mouvements de la rue, celui de conduire à la paralysie et à l'abandon des réformes, et, peut-être, à pire encore. Or, nous le savons tous, notre pays a besoin de réformes ; malheureusement, plus nous avançons dans le quinquennat, plus les réformes structurelles s'éloignent. J'en viens au projet de loi de financement de la sécurité sociale tel qu'il a été modifié par les députés et le Gouvernement. Je fais trois constats

Premier constat : la non-compensation par l'État des recettes supprimées du fait des mesures prises en réponse au mouvement des « gilets jaunes » est confirmée. Nous pensons que cette disposition marque une rupture dans le pacte d'autonomie de la sécurité sociale. L'instauration de ce que j'appelle la « bercysation » du financement de la sécurité sociale est une atteinte directe à notre modèle social. Exact ! En effet, le principe fondateur de notre protection sociale, en vertu duquel « chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins », reste parfaitement d'actualité. Nous le voyons bien, ces milliards d'euros manquent cruellement au budget de la sécurité sociale, au moment même où il serait nécessaire de donner un nouveau souffle à l'hôpital- j'y reviendrai dans quelques instants. Deuxième constat : cette situation de « déficit organisé » par le Gouvernement entraîne le maintien plus que contestable d'un plan d'austérité ... Très juste ! Vous Je pense tout d'abord à la non-revalorisation des pensions à hauteur de l'inflation, qui va avoir pour effet une nouvelle baisse du pouvoir d'achat pour une partie des retraités. Cette mesure est d'autant plus critiquable qu'elle s'avère fragile vue du principe constitutionnel d'égalité, comme l'a souligné notre collègue René-Paul Savary dans son rapport. Elle permet en effet à un assuré dont les revenus du capital sont importants mais la pension faible de bénéficier d'une revalorisation au niveau de l'inflation, alors qu'un autre assuré, dont les revenus globaux peuvent être moins importants mais dont la pension est supérieure à 2 000 euros, ne voit sa pension revalorisée que de 0,3 %. Nous pensons donc que la question se pose, au regard du principe contributif, de Par ailleurs, la confirmation de la sous-indexation des prestations familiales met une nouvelle fois à mal la politique familiale. Alors que la situation financière de la branche s'est améliorée depuis 2018, il est injuste que les familles subissent davantage de mesures pénalisantes pour leur pouvoir d'achat. Je vous rappelle, mes chers collègues, que, depuis 2014, les familles ont subi : la modulation des allocations familiales, dont l'effet cumulé, depuis cette date, s'élève à 3,4 milliards d'euros la suppression du complément de libre choix d'activité majoré, qui représente 490 millions d'euros non perçus entre 2014 et 2019 ; la modulation de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE), dont l'effet cumulé, toujours depuis 2014, s'élève à 870 millions d'euros ; l'alignement du montant et du plafond de l'allocation de base sur le complément familial, qui représente 260 millions d'euros entre 2018 et 2019. L'accumulation de ces mesures fait perdre à la branche famille son rôle essentiel de compensation des charges de famille. Certes, le gouvernement actuel n'est pas à l'origine de toutes ces mesures, mais il n'a pas renoncé à l'héritage et n'a fait que poursuivre la casse de la politique familiale. La majorité sénatoriale ne cesse de le rappeler : il est temps de mettre fin à ces mesures d'économies faites sur le dos des familles. Comme le souligne notre collègue Élisabeth Doineau dans son rapport, il est temps de reconstruire les moyens de relancer une politique familiale ambitieuse. Eu égard notamment à la baisse de 8,5 % en dix ans du nombre de naissances, il nous semble indispensable de changer de politique dans ce domaine. Concernant le secteur de la santé- notre collègue Catherine Deroche l'a très bien dit en première lecture -, si nous reconnaissons, dans ce PLFSS, des avancées que nous soutiendrons, ce texte nous laisse cependant un goût d'inachevé au regard des enjeux inédits auxquels fait face notre système de santé. Nous considérons que la réponse donnée à la crise de l'hôpital n'est pas à la hauteur des enjeux. Depuis six mois, que fait le Gouvernement pour l'hôpital ? Il va de plan d'urgence en plan d'urgence : un premier plan pour les urgences, en juin dernier, et, à la clé, 70 millions d'euros sous forme de primes ; puis, en septembre, un nouveau plan, à 750 millions d'euros cette fois, mais sur trois ans, ces deux plans deux plans étant financés par un redéploiement de crédits. Vient enfin un troisième plan de « soutien ». Cette fois, le montant annoncé est de 1,5 milliard d'euros sur trois ans, mais seulement 300 millions d'euros pour 2020.

Quant à la reprise du tiers de la dette des hôpitaux, elle doit permettre à ces derniers de réduire leur déficit et de retrouver rapidement les moyens d'investir. Mais qui décidera de ces investissements ? Les professionnels de santé attendaient un plan de sauvetage. Or les revalorisations se sont transformées en primes ponctuelles, soumises à conditions. Qui plus est, ces primes ne seront pas destinées à l'ensemble des personnels hospitaliers : certaines d'entre elles ne concerneront que les personnels de quelques départements franciliens. Nous estimons qu'opposer les territoires n'est pas une bonne politique. À passer le budget des hôpitaux sous la toise, à grand renfort de mesures de régulation censées nous permettre de tenir l'Ondam, tout le système craque. Il faut réarmer l'hôpital ! Le Gouvernement ne fait pas complètement ce choix. À long terme, nous savons que les besoins de financement des hôpitaux vont s'accroître, car ceux-ci sont confrontés à une hausse structurelle de leurs dépenses, liée à l'évolution démographique, au vieillissement et à l'innovation médicale, ainsi qu'aux attentes des patients. Nous ne pouvons donc pas considérer les annonces faites par le Premier ministre comme des mesures d'ampleur ; elles n'ont d'ailleurs pas rassuré les professionnels de santé. Nous considérons désormais que, sans une réforme systémique, les PLFSS se suivront à l'identique au désespoir des soignants et des soignés.

et rendre le pouvoir à ceux qui soignent. Réformer, c'est aussi accepter de donner une juste rémunération aux personnels pour rendre réellement les métiers attractifs. C'est également régionaliser l'organisation de la santé pour y impliquer les collectivités locales et se rapprocher des besoins de terrain. Je terminerai mon intervention par un troisième constat : ce PLFSS traduit l'inaction du Gouvernement par rapport au déficit des régimes de retraite. Or il faut agir sans attendre une réforme systémique qui, peut-être, ne viendra pas. Au motif de l'injustice des régimes spéciaux, le Gouvernement s'est lancé dans une vaste entreprise qui pourrait conduire à réformer tout le reste, en laissant de côté ces mêmes régimes qui ne rentreraient qu'un jour peut-être dans le système universel. Ces derniers jours, le Gouvernement a renoncé à la fameuse « clause du grand-père », au profit d'une adaptation de la réforme des retraites « secteur par secteur ». Cela revient donc à conserver les inégalités qu'il s'agissait de supprimer En outre, alors que ce PLFSS présente une forte dégradation du solde de la branche vieillesse pour la période 2020-2023, la seule réponse proposée, cette année encore, est de sous-revaloriser les pensions. Depuis plusieurs années, la majorité sénatoriale plaide pour un relèvement progressif de l'âge minimum légal de la retraite, seul à même de rétablir une trajectoire financière positive pour la décennie 2020. Si rien n'est fait, les retraités actuels continueront à voir leur pension diminuer et les futurs retraités auront des retraites beaucoup plus faibles. Exact ! Cette paupérisation des retraités, nous n'en voulons pas Nous pensons que les Français sont prêts à entendre un discours de vérité. En revanche, la cacophonie gouvernementale actuelle ne fait que les angoisser. le groupe Les Républicains adoptera un texte amendé en vue de donner plus de pouvoir d'achat aux retraités et aux familles et s'opposera à l'Ondam, qu'il considère sous-dimensionné par rapport aux besoins de l'hôpital. Bravo

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, où en sommes-nous aujourd'hui de la déstructuration de la sécurité sociale ? L'automne 2018 annonçait un hiver 2019-2020 plein d'espoir fondé sur un équilibre retrouvé. Même si l'ombre de Bercy planait sur les excédents à venir, les plus optimistes rêvaient de crédits nouveaux renforçant le plan Ma santé 2022, apportant des remèdes solides à la crise de l'hôpital public, amorçant une grande loi de l'autonomie. À l'automne 2019, une révolte sociale non maîtrisée, une conjoncture moins favorable qu'envisagé et surtout des choix politiques assumant une vision régressive de la sécurité sociale conduisent à un projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 qui creuse ce que j'appellerai un nouveau « trou politique » de la sécurité sociale, qui abaisse le pouvoir d'achat des familles et d'une partie des retraités, qui ignore, sinon méprise, les forces intermédiaires de la démocratie, syndicales et parlementaires, provoquant dans notre chambre haute un véritable gâchis- l'arrêt de l'examen des articles

J'insisterai sur deux points. Premièrement, la non-compensation des exonérations de cotisations par le budget de l'État n'est pas un simple acte technique. Comment

dans la baisse des recettes, qu'amplifie le transfert du financement de deux agences nationales, le moyen de forcer celle des dépenses ? Plus grave est la rupture du contrat social de 1944, qui marque un changement complet de philosophie de la « sécu ». Celle-ci ne doit pas, je l'ai souvent souligné, évoluer vers une institution à l'anglo-saxonne d'assistance aux plus défavorisés. Cela détruirait un pilier de solidarisation de la société et tarirait une source de démocratie sociale. Deuxièmement, la détermination des collectifs Inter-Blocs, Inter-Urgences et Inter-Hôpitaux, des associations, des organisations syndicales médicales et paramédicales à poursuivre ensemble leur mobilisation ce samedi manifeste la forte déception ressentie le 17 novembre. En effet, les revalorisations salariales sont très en deçà des attentes, avec une distribution de primes- surtout franciliennes -sans augmentation du point d'indice, alors que c'était l'une des principales revendications des infirmiers et aides-soignantes, dont les salaires sont parmi les plus bas de l'Union européenne. outre, il n'y a pas de volonté affirmée de mettre fin aux fermetures de lits. En une vingtaine d'années, 100 000 lits ont été supprimés, au grand dam des urgentistes, qui dénoncent le manque de places pour hospitaliser leurs patients.

Il est urgent de poser la question de la place de l'hôpital, de ses missions, des valeurs et du sens que nous souhaitons voir inspirer notre système public hospitalier quand la médecine connaît des bouleversements majeurs. en ces termes dans notre hémicycle, le 8 juin 1994 : « Gardons-nous d'oublier notre bien commun qu'est la sécurité sociale ! Gardons-nous de l'appréhender seulement sous l'angle des charges et des déficits ! La sécurité sociale, [ ...] c'est d'abord un immense progrès social et le plus puissant facteur de cohésion sociale qui existe en France et que nous avons le devoir de préserver pour les générations futures. » Pour conclure, je laisse la parole à une

d'un nouveau fonds d'indemnisation pour les victimes de maladies liées aux pesticides ou encore d'un service public de versement des pensions alimentaires. Par ailleurs, 500 millions d'euros seront dégagés pour le grand âge et l'autonomie.

vous avez annoncé 1,5 milliard d'euros supplémentaires sur trois ans, la reprise du tiers de la dette de l'hôpital, à hauteur de 10 milliards d'euros, et une série de primes nouvelles pour certains soignants. S'agissant de la reprise de la dette, qui a été bien reçue par les établissements, des interrogations persistent, en particulier concernant les hôpitaux qui vont en bénéficier. Cette reprise partielle ne risque-t-elle pas de remplacer certaines subventions aux opérations d'investissement ? Un éclaircissement sur ce point, madame la ministre, serait le bienvenu. Ce plan, complété par la pluriannualité des financements, tant attendue par les professionnels, est salué par les établissements hospitaliers publics, qui retrouvent des marges de manoeuvre permettant d'améliorer le quotidien des soignants et des patients. On doit le saluer Toutefois, une incompréhension a émergé au sein des établissements privés à but non lucratif, qui assument pour la plupart des missions de service public. Sur certains territoires éloignés des CHU, ils peuvent même être les seuls établissements à proposer une offre de soins et à la structurer. Comme leurs homologues du secteur public, ils font face à des baisses considérables de tarifs depuis de trop nombreuses années, tout en supportant des charges plus élevées : par exemple, une prime de 100 euros au personnel coûte 146 euros à l'hôpital public, contre 201 euros Madame la ministre, ces nouvelles mesures n'auraient-elles pas pu profiter à toutes les filières de soins qui concourent à une mission d'intérêt général ?

notamment en ce qui concerne les professions paramédicales. Quand le salaire d'une infirmière est en France de 1 700 euros, il est de 3 200 euros au Luxembourg, à ancienneté et à compétence égales. Ainsi, les professionnels que nous formons en France sont aspirés par les pays voisins.

aujourd'hui, faute d'application uniforme du décret, les établissements ayant tenté de s'y conformer s'en sont trouvés pénalisés. Au CHRU de Nancy, par exemple, dans la semaine suivant le début de l'application du décret, plus aucun intérimaire n'a accepté de revenir

de santé, qui demandent rigueur et exigence et dont nous avons tant besoin. La revalorisation par prime est la bienvenue, mais elle ne devrait être qu'une étape vers la revalorisation des salaires.

Qui pourrait affirmer pouvoir remédier, au travers d'un seul budget, à des décennies d'errements, de manque d'anticipation, à des années de tarification à l'activité, de baisse des tarifs et de non-revalorisation des salaires ?

nouvelle lecture du PLFSS pour 2020 se déroule dans un contexte un peu particulier. Alors que le Président de la République s'exprimait à Épernay sur la problématique de l'hôpital, notre chambre a brutalement décidé d'abréger, jeudi 14 novembre, la discussion du texte, protestant contre ce qu'une partie de ses membres considérait être une marque de « mépris » de l'exécutif envers le Parlement. C'était du mépris ! Mes chers collègues, que fallait-il faire ? La situation actuelle est un bien triste héritage. Depuis plus de quinze ans, plusieurs réformes ont profondément affecté le personnel en charge des patients droits des malades, réforme de simplification, grands plans pour les hôpitaux, loi de modernisation de 2016 ... Et je ne parle pas de l'application des 35 heures sans contrepartie ! Un malaise s'est installé chez l'ensemble des personnels hospitaliers : leur ras-le-bol s'est exprimé cette année. Mes chers collègues, que fallait-il faire ? Ignorer la pression budgétaire à laquelle l'hôpital public doit faire face depuis des années ? Ignorer le malaise qui couvait à l'hôpital public et qui a pris ces derniers mois une ampleur nouvelle ? Masquer le déficit d'investissement qui oblige à une vision court-termiste ? Négliger le personnel ? Nous lui devons tellement .... Nous avons eu l'occasion de dire les difficultés que connaît l'hôpital public, et nous admettons tous Pour y répondre, les nécessaires mesures structurantes ont été prises avec la stratégie Ma santé 2022. Cependant, les dernières mobilisations ont montré l'épuisement, voire la colère, de ceux qui travaillent quotidiennement Répondre à l'important ne suffisait pas ; il fallait répondre à l'urgent immédiatement. Le Président de la République, reprenant vos propos, madame la ministre, a rappelé que nous devions entendre les besoins exprimés par les personnels hospitaliers, afin d'accompagner leurs efforts et de poursuivre la transformation. À Épernay, il vous a demandé formellement d'en accélérer la mise en oeuvre, sous l'autorité du Premier ministre. Présentées la semaine passée, les conclusions de ces travaux comportent une série de mesures visant à investir dans l'hôpital et à soutenir la transformation engagée par le plan Ma santé 2022.

une meilleure revalorisation- les aides-soignants, par exemple, auront des possibilités d'accéder à la catégorie B de la fonction publique en fin de carrière -ou par le versement de trois sortes de primes une prime territoriale de 800 euros, attribuée aux personnels hospitaliers de la région parisienne, où recruter est un souci majeur ; une prime sectorielle pour le personnel hospitalier qui exerce dans les services de gériatrie ; une prime managériale de 300 euros en moyenne par personne et par an, réservée à des personnels qui s'investiront dans des actes spécifiques. Deuxièmement, il faut « remettre tous les soignants, médecins, infirmiers, aides-soignants au coeur de la gouvernance des hôpitaux Pour accélérer la transformation entreprise avec le plan Ma santé 2022, vous avez proposé, madame la ministre, de renforcer et de valoriser le management de proximité. Par exemple, les médecins pourront devenir directeurs d'hôpital. Vous proposez également de simplifier le fonctionnement, par exemple pour les formalités de recrutement ou les protocoles de coopération décentralisés. Troisièmement, il faut « réinvestir l'hôpital public en lui donnant des moyens nouveaux et de la visibilité dans le temps mesures. Tout d'abord, la hausse des tarifs hospitaliers d'au moins 0,2 % par an jusqu'à la fin du quinquennat : pour rappel, mes chers collègues, l'inversion de la courbe s'est faite en 2019, mettant fin à dix années de baisses successives. d'investissement courant ensuite, les hôpitaux pourront acheter le matériel indispensable pour le travail des soignants au quotidien. Enfin, s'agissant de l'investissement à long terme, la reprise d'un tiers de la dette des hôpitaux, soit 10 milliards

Cet effort supplémentaire atteindra 1,5 milliard d'euros à la fin du quinquennat. Elles ont également eu pour effet de flécher 150 millions vers l'investissement courant en 2020, afin de répondre aux besoins actuels les plus forts. Cet effort sera reconduit en 2021 et en 2022. enfin entraîné une révision des tableaux récapitulatifs pour 2020 et une adaptation de la trajectoire quadriennale de la sécurité sociale. Ces ajouts viennent conforter le texte présenté à notre chambre il y a trois semaines et dont je me dois de rappeler les mesures phares, qui répondent à un double objectif de réduction des impôts et de justice sociale. Le PLFSS est axé sur la récompense du travail, avec la poursuite de l'exonération de cotisations sociales sur les heures supplémentaires, la protection des plus fragiles, avec la pérennisation de la revalorisation de la prime d'activité à hauteur de plus de 90 euros en janvier 2019 et la revalorisation de l'AAH et du minimum vieillesse, la lutte contre la perte d'autonomie, au travers de l'article 45, qui met en place un congé indemnisé de proche aidant, la lutte contre les inégalités de destin, au travers par exemple de l'article 40, qui prévoit le remboursement d'un forfait pour l'accompagnement des patients après un cancer, l'amélioration des prises en charge et de l'accès aux soins dans tous les territoires. Je pense notamment, à cet égard, à l'article 37, qui vise à mettre en oeuvre un forfait transport-hébergement pour les femmes enceintes résidant à plus de quarante-cinq minutes d'une maternité. Voilà, mes chers collègues, quelques-unes des grandes avancées de ce PLFSS pour 2020. C'est un texte qui trace des perspectives d'avenir, qui montre la voie du progrès social, qui rétablit la justice sociale, qui investit dans le système de santé au bénéfice des patients et du personnel soignant, qui répond à l'urgence sans remettre en cause l'important. Et qui guérit

Ces tensions se faisaient ressentir au second trimestre de cette année, c'est-à-dire au moment où le Gouvernement commençait à penser les grands équilibres du PLFSS. Or force est de constater que, malgré cette crise, le Gouvernement construisait un sous-Ondam hospitalier inférieur au sous-Ondam de ville. Dès lors, ce PLFSS ne pouvait ni apaiser les professionnels hospitaliers ni rassurer les parlementaires, singulièrement les sénateurs, qui alertaient depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Reconnaissons qu'entre-temps le Gouvernement n'est pas resté sans agir : il a proposé, en juin, 70 millions d'euros pour les urgences, puis, en septembre, 750 millions d'euros pour tout l'hôpital. Malheureusement, cela s'est avéré insuffisant pour remédier à la situation. S'il faut saluer la réponse du Président de la République aux manifestations, il est regrettable que l'entière mesure de la situation n'ait pas été prise préalablement. En effet, cela a obligé le Gouvernement à réévaluer l'Ondam pendant l'examen au Sénat du PLFSS, tout en nous demandant d'adopter un texte manifestement insincère. C'est la raison pour laquelle nous étions dans notre bon droit en rejetant ce texte il y a deux semaines. Aujourd'hui, nous sommes absolument dans notre rôle, et nous ne pouvions pas nous soustraire à l'examen du budget de la sécurité sociale, qui représente 522,1 milliards d'euros, en adoptant une motion tendant Évidemment, les règles constitutionnelles, en particulier celle de l'entonnoir, limitent à ce stade de la procédure notre pouvoir d'amendement. Mais je ne doute pas, mes chers collègues, que le texte que nous adopterons portera la marque du Sénat et comportera quelques mesures symboliques sur lesquelles J'espère, madame la ministre, que, en raison de ces conditions d'examen très particulières, l'Assemblée nationale saura redoubler d'attention lorsqu'elle aura à se prononcer en dernier ressort sur les amendements que nous aurons adoptés. Nous comptons sur votre compréhension et sur votre bienveillance.

Or cette doctrine s'appuie sur un simple rapport rendu au Gouvernement il y a un an par MM. Charpy et Dubertret. Vous conviendrez, mes chers collègues, qu'il apparaît inopportun, voire déplacé, de soutenir devant le législateur la suprématie d'un rapport sur la loi elle-même

Le PLFSS initial comportait un sous-Ondam hospitalier inférieur au sous-Ondam de ville, alors que nos services des urgences et nos hôpitaux sont en grève depuis de longs mois : cela constituait un premier motif d'incompréhension. S'ajoutait le fait que l'Ondam était présenté comme étant à la hausse : cela est vrai, mais les professionnels du secteur, parfois épuisés, relevaient surtout que, même en progression, il restait bien inférieur à l'évolution tendancielle des dépenses.

Rappelons-nous, mes chers collègues, qu'avant la création de l'Ondam notre système n'était plus tenable. Aujourd'hui, on constate durement que la gestion par l'Ondam ne peut, à elle seule, suffire au pilotage de notre système. Nous ne pourrons pas faire abstraction du constat énoncé par collègue Olivier Henno en première lecture : « Reporter les coûts de notre santé et de notre sécurité sociale sur d'autres générations et les financer par l'emprunt apparaîtront comme une aberration. Sans modification profonde de notre système de santé, limiter la progression l'Ondam implique l'endettement direct des hôpitaux. Le Premier ministre, à l'occasion de la présentation du plan Hôpital, rappelait que l'investissement hospitalier a été divisé par deux en dix ans, alors que la dette des hôpitaux augmentait de 40 %. Un ouvrage profond et difficile est sur le métier : il est primordial de revoir la gouvernance de l'hôpital, de favoriser l'ambulatoire et de réorienter notre médecine vers la prévention ; il est fondamental de regarder ce qui se pratique hors de nos frontières, un récent rapport de l'OCDE pointant les grands gagnants parmi les systèmes de santé dans le monde. certainement de sources d'inspiration importantes, qui pourront guider les réflexions demandées par le Gouvernement. Toutefois, dans l'immédiat, nos équipes soignantes attendent des réponses massives. Si l'on peut reconnaître au Gouvernement le mérite de ne pas retenir l'option du redéploiement de moyens, on peut s'interroger sur les annonces.

Concernant les revalorisations à hauteur de 0,3 % plutôt qu'au niveau de l'inflation des pensions de retraite et des prestations sociales, ce procédé semble devenir un levier d'économie classique pour le Gouvernement ; nous le regrettons, et nous soutiendrons l'amendement de notre rapporteur Concernant le dispositif relatif aux assistantes maternelles, nous nous réjouissons que la proposition de notre collègue rapporteur Élisabeth Doineau ait été reprise purement et simplement par l'Assemblée nationale. Concernant le fractionnement du congé de présence parental, j'avais proposé en première lecture de l'étendre aux trois fonctions publiques. Je me félicite que les députés aient adopté

les sénateurs du groupe socialiste et républicain ont déploré que le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, tel que présenté en première lecture, ne soit ni réaliste ni sincère et qu'il ne permette pas de répondre aux enjeux et aux besoins, en particulier ceux de l'hôpital. Faute d'être entendus, suspendus à une éventuelle réaction gouvernementale, à une intervention présidentielle, nous avons été contraints de mettre fin à ce qui s'apparentait à une mascarade de débat, et donc de rejeter ce texte. Cette séquence très particulière a permis d'illustrer, une fois de plus, le manque de considération du Gouvernement non pas uniquement pour le Sénat, mais pour le Parlement dans son ensemble. Aujourd'hui, nous avons tous l'impression désagréable de revivre la même situation que l'an dernier, lorsque l'exécutif avait opéré un revirement de dernière minute et cédé à des demandes que nous faisions nous-mêmes depuis plusieurs mois ; je pense notamment à l'exonération de l'augmentation de la CSG pour les retraités modestes. Cette année, nous vous avons alertés à plusieurs reprises sur les dangers de la cure d'austérité imposée aux hôpitaux. En vain ... Et nous nous retrouvons donc ce week-end pour débattre de mesures présentées par le Gouvernement en urgence, quelques jours après la grande mobilisation du 14 novembre visant à défendre l'hôpital public et notre système de santé et huit mois après le début de la grève des services des urgences

750 millions d'euros, on se perd dans les chiffres ! -, déjà totalement déconnectées et insuffisantes pour sauver l'hôpital. Nous souhaiterions, au-delà de toutes ces communications successives, parler des vrais sujets les retards d'investissement, la dégradation des conditions de travail et de prise en charge des patients, les sous-effectifs et les problèmes de sécurité dans les services, le manque de lits, la sous-rémunération des personnels soignants ... Oui, revenons-en au fond de ce plan prétendument « sans précédent », « historique

aux primes pour les soignants, il n'y en aura de toute évidence pas pour tout le monde. Primes pour les uns, mais pas pour les autres, sous prétexte qu'ils ne sont pas franciliens : vous opposez Paris aux déserts médicaux français ! À cet instant, toutes mes pensées vont aux personnels, et plus particulièrement aux infirmiers et aux aides-soignants, des hôpitaux de

que vos propositions ne répondent pas aux attentes en matière de reconnaissance du travail, des métiers ou de la pénibilité des tâches, et plus globalement au problème du manque d'attractivité des hôpitaux. Je rappelle que la première revendication de ces personnels est d'être suffisamment nombreux pour pratiquer les soins, pour être en mesure de faire convenablement leur travail, de sauver des vies. Or, au final, trop de questions restent sans réponse : des embauches, de l'arrêt des fermetures de lits, de l'organisation territoriale des soins ou encore de la prise en charge spécifique de la perte d'autonomie ? Rien, il n'y a rien de précis,

On l'aura compris, cette nouvelle version du texte n'est pas beaucoup plus réaliste que la première et, d'après ce que j'ai pu observer, il n'est pas de nature à faire retomber la mobilisation sociale. Décevant, il risque surtout d'attiser la colère. Il ne serait donc pas responsable d'en rester là.

», en violation de la loi Veil de 1994. Les cotisations sociales des Français servent notamment à garantir leur retraite et à assurer leur santé, non à pallier votre politique budgétaire défaillante. Comme il y a quinze jours, nous sommes en désaccord profond avec toutes les mesures tendant à réduire le pouvoir d'achat des Français ; je pense en particulier à la désindexation de certaines retraites et prestations sociales. Le budget de la sécurité sociale traduit le niveau des droits sociaux que la Nation accorde à ses concitoyens pour faire face aux aléas de l'existence. Le projet de loi de finances pour 2020, s'il est voté en l'état, ne dérogera pas aux deux précédents : il affaiblira notre système de santé et creusera les inégalités. est la réalité, et nous nous battrons, durant les deux jours à venir, pour faire valoir notre vision du pacte social républicain, différente de la vôtre.

peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt assis sur les rémunérations qu'ils versent à leurs salariés au cours de l'année civile L'article 3 du PLFSS pour 2020 prévoit, quant à lui, que ce crédit d'impôt ne fasse pas l'objet d'une compensation à la sécurité sociale. Or les compensations de pertes de recettes ou de transferts de charges entre l'État et la sécurité sociale sont régies par le principe de « compensation intégrale » défini à l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. De plus, cette politique d'exonération de cotisations sociales a des conséquences directes sur le financement de notre système de protection sociale, fondé sur la solidarité Par ailleurs, la Cour des comptes relève, dans son dernier rapport, un déséquilibre des comptes de la sécurité sociale qui s'explique, avant tout, par la politique d'exonération de cotisations sociales. C'est la raison pour laquelle est proposée la suppression de cet article.

qui n'a fait l'objet d'aucune approbation par le Parlement. Ce rapport préconise de revenir sur la règle de la compensation intégrale relative aux allégements généraux, lesquels, rappelons-le, représentent au total 66 milliards d'euros pour 2019. On voit bien jusqu'où peut conduire cette logique de la non-compensation d'un très gros manque à gagner- et à dépenser -pour la sécurité sociale, dont nous avons tous rappelé les immenses besoins. Le système de tuyauterie entre le budget de l'État et celui de la sécurité sociale est devenu extrêmement complexe, mais l'argent coule toujours dans le même sens, de la sécurité sociale vers l'État, et beaucoup plus rarement dans l'autre sens. Pour ces raisons nous demandons la suppression de l'article 3. Quel

En outre, 5,1 milliards d'euros du budget général sont affectés à la compensation à l'euro près des exonérations ciblées, puisque les mesures non compensées concernent la suppression d'une disposition relative à la modulation du taux de CSG et l'exonération de cotisations sociales

Les compensations de pertes de recettes ou de transferts de charges entre l'État et la sécurité sociale sont pourtant régies par le principe de « compensation intégrale Depuis 2017, des entorses à cette règle ont été observées. Par exemple, le crédit d'impôt sur la taxe sur les salaires (CITS) n'a pas fait l'objet d'une compensation à la sécurité sociale en 2018. de recettes non compensées à la sécurité sociale s'élèveraient à un montant estimé à 3,5 milliards d'euros : 1,2 milliard d'euros d'exonération de cotisations sociales sur les heures supplémentaires, 1,5 milliard d'euros de baisse de la CSG pour les retraités gagnant moins de 2 000 euros par mois et une diminution de 800 millions d'euros du forfait social. Par conséquent, l'article 3 prive la sécurité sociale de 3,5 milliards d'euros de ressources qui devraient lui revenir, ce qui n'est pas acceptable. C'est pourquoi le présent amendement vise à supprimer les alinéas de l'article relatifs à cette non-compensation.

de quoi il s'agit. L'article 3 du PLFSS prévoit que les pertes de recettes résultant de l'avancement au 1 janvier 2019 de l'exonération de cotisations sociales

Ces deux mesures représentent une perte de recettes de près de 3 milliards d'euros en 2019 pour la sécurité sociale, ce qui explique en grande partie le retournement de situation financière et la reprise de la dégradation des comptes sociaux.

opposés à cette rupture avec la loi de 1994, non par nostalgie d'un passé idéalisé, mais parce que cette doctrine que cette doctrine nouvelle affirmée et mise en oeuvre par le Gouvernement est destructrice, à nos yeux, du pacte de la sécurité sociale, fondé sur la solidarité des bien-portants avec les malades,

prévoit actuellement un plan social de 300 personnes, malgré un bénéfice net de 6 milliards d'euros en 2018 ! En outre, ces entreprises continuent malgré tout d'engranger de l'argent public

de ponctionner les caisses de la sécurité sociale pour augmenter les bénéfices du secteur privé ! Doit-on vous rappeler, monsieur le secrétaire d'État, que les industries pharmaceutiques ne sont pas des entreprises publiques et que les bénéfices qu'elles dégagent vont directement dans les poches de leurs actionnaires ?

À mon sens, la possibilité de fixer annuellement ce seuil de déclenchement constitue, pour le législateur, un moyen simple et transparent de redéfinir l'assiette de l'impôt au regard des capacités contributives des entreprises imposables. Il me semble tout à fait opportun

Or les mesures contenues dans le présent PLFSS ne sont pas à la mesure des enjeux. Les dépenses en faveur des établissements de santé sont tout particulièrement insuffisantes, à l'heure où l'hôpital public est en très grande difficulté. Le Gouvernement promettait, lors de l'examen du plan Ma santé 2022, de renforcer les hôpitaux de proximité. Un tel Ondam rend impossible la tenue de telles promesses, puisque les moyens alloués sont complètement sous-évalués.

Il est à craindre, en effet, que les salariés des petites entreprises ne soient exclus, une fois de plus, d'un dispositif de soutien au pouvoir d'achat. Une telle restriction ne paraît pas juste. L'amendement

Maurice Antiste. Cet amendement vise à permettre aux entreprises de gratifier, si elles en ont la possibilité, leurs collaborateurs sans devoir payer de charges patronales. Cette mesure doit également pouvoir être reconduite d'une année sur l'autre. Elle constituera ainsi un moyen de soutenir le pouvoir d'achat des ménages, mais aussi de valoriser le travail des salariés.

donc émis un avis défavorable

Nous proposons de supprimer les dispositions de l'article relatives au bonus-malus sur les cotisations patronales d'assurance chômage en fonction de l'utilisation de contrats courts par les employeurs.

patronales sur les bas salaires, dites « réductions Fillon ». Ces exonérations et allégements ne font que maintenir les salariés dans la précarité, avec des salaires ne dépassant pas 1,4 fois le SMIC : au-delà, les employeurs ne bénéficient plus des exonérations et allégements, ce qui crée un effet d'aubaine. Ce dispositif n'améliore en rien la situation de l'emploi, car, contrairement à ce qu'a affirmé le rapporteur général lors de la première lecture, la France connaît toujours aujourd'hui un chômage de masse. Permettez-nous d'adopter un regard critique sur des évaluations de politiques publiques faites par des organismes

Monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, nous ne pouvons plus accompagner les entreprises dans leur chantage à l'emploi, qui prive les travailleurs et travailleuses de ce pays de conditions de travail et de vie dignes, ainsi que d'une protection sociale de qualité

particulièrement performants à plus de 120 millions d'euros. Le Gouvernement, quant à lui, a reconnu une ponction de 66 millions d'euros, voire de 70 millions d'euros, sur les entreprises ultramarines.

dont le coût pour la sécurité sociale n'est pas compensé par l'État. Ainsi, la sécurité sociale est doublement perdante : elle perd à la fois le produit des cotisations sociales sur les indemnités de rupture conventionnelle et les cotisations sociales dues au titre d'une relation de travail pérenne. constater, monsieur le président, que j'ai défendu deux amendements en un temps record ; le chronomètre ne s'est même pas déclenché !